L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'énergie et au climat

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en juillet dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'énergie et au climat a été conclusive. Je me félicite que le Sénat et l'Assemblée nationale soient convenus d'un texte de compromis sur un sujet aussi essentiel, un texte qui concourra à atteindre l'objectif de neutralité carbone issu de l'accord de Paris de 2015.

Je salue également ma collègue Pascale Bories, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, pour la qualité du dialogue entre nos commissions. Au terme de son examen, le texte, qualifié de « petite loi énergie » au sortir du conseil des ministres, comporte soixante-neuf articles, contre douze initialement.

Face à l'urgence climatique, je crois que le Sénat a pleinement joué son rôle pour rehausser sensiblement ce niveau d'ambition. Pour autant, le Gouvernement aurait pu faire davantage en matière de soutien aux entreprises, notamment les plus consommatrices d'énergie,

La commission des affaires économiques, dont je remercie la présidente, Sophie Primas, et tous les autres membres, a donc su faire progresser sa vision singulière des conditions de réussite de la transition énergétique. Nous en sommes convaincus : cette transition ne pourra aboutir que soutenue par des objectifs ambitieux et crédibles de diversification de notre mix, qui doivent être déterminés par le Parlement et non par un cénacle d'experts elle requiert des normes aussi simples que possible, qui privilégient la confiance plutôt que la contrainte, l'incitation économique plutôt que l'alourdissement fiscal, le droit souple plutôt que l'étouffement normatif elle repose avant tout sur des actions décentralisées, mises en oeuvre par nos entreprises et nos collectivités territoriales, mais aussi par les citoyens, autour d'un État facilitateur, garant de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires horizon partagé la promotion de nouveaux modes de production et de consommation plutôt que le renoncement à la croissance économique et,, au progrès social. C'est dans cet esprit que nous nous sommes efforcés d'infléchir et d'enrichir le texte, en agissant dans quatre directions. En premier lieu, le Sénat a notablement relevé les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d'adresser un signal fort en direction de la structuration des filières de l'économie verte. C'est sur son initiative qu'ont été inscrites dans le code de l'énergie des orientations visant notamment à encourager la petite hydroélectricité, à porter le rythme d'attribution des appels d'offres pour l'éolien en mer à 1 gigawatt par an d'ici à 2024, à atteindre 20 à 40 % d'hydrogène vert dans la consommation totale d'hydrogène en 2030 et à valoriser la biomasse à des fins de production d'énergie, en maintenant la priorité donnée à la production alimentaire. Ces objectifs offriront aux acteurs économiques la visibilité qu'ils sont en droit d'attendre. En deuxième lieu, le Sénat a substantiellement renforcé la loi quinquennale qui déterminera, dès 2023, notre politique énergétique. En particulier, il a étendu le périmètre

variant de 10 à 60 %. Dans le même ordre d'idées, le Sénat a prévu la fixation par cette loi des volumes maximal et minimal des certificats d'économies d'énergie, les CEE. Il s'agit d'une avancée majeure pour le Parlement, mais aussi pour les consommateurs, puisque ces concentrent un volume financier de plus de 3 milliards d'euros, soit 3 à 4 % de la facture d'énergie. Convaincu de la nécessité d'inverser la hiérarchie des normes en matière énergétique, le Sénat a établi la primauté de la loi quinquennale sur les autres documents de planification, à commencer par la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, et la stratégie nationale bas-carbone. Face aux changements climatiques, qui posent aussi un défi démocratique, il a ainsi voulu affirmer la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire, de la politique sur la technique. dernier apport notable à la loi quinquennale consiste en l'évaluation dont elle fera l'objet lors de chaque projet de loi de finances initiale. En complétant ainsi l'information budgétaire des parlementaires, notre assemblée a souhaité que les orientations fixées par la loi, qui ne sauraient rester déclamatoires, puissent être déclinées

Dans le même esprit, il a assoupli les conditions de mise en oeuvre des projets d'autoconsommation par les organismes d'HLM. En dernier lieu, notre assemblée a veillé à accompagner l'ensemble des parties prenantes, des entreprises aux collectivités territoriales, une préoccupation qui l'a d'abord conduite à adopter des mesures d'accompagnement pour les salariés touchés par la fermeture des centrales à charbon. Le Sénat a aussi cherché à consolider les ressources d'EDF, tout en préservant un coût compétitif pour les consommateurs, en prévoyant que le prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, l'Arenh, pourra être révisé en fonction de l'inflation. Il appartiendra au Gouvernement de fixer par voie réglementaire un prix et un niveau d'Arenh adéquats, dans le respect de trois exigences : une juste rémunération du parc nucléaire et la possibilité de disposer d'offres alternatives, mais, avant tout, un prix bon marché pour les consommateurs. Au-delà de cette mesure ponctuelle, la commission des affaires économiques sera très attentive au projet de réorganisation d'EDF, opportunément dénommé « Hercule », étant donné l'ampleur de l'objectif visé, mais aussi de l'inquiétude suscitée. Plus largement, notre commission fera preuve d'une grande vigilance sur l'évolution de la filière nucléaire, à l'heure où l'abandon du projet de réacteur de quatrième génération, Astrid, fait augurer une baisse regrettable de notre ambition scientifique dans ce domaine.

S'agissant des collectivités territoriales, le texte offre aux élus locaux, notamment aux maires, une boîte à outils qui leur sera très utile pour faire de la transition énergétique un levier de développement local au coeur de nos territoires. Par exemple, les communes pourront financer leurs travaux de rénovation avec des CEE, contribuer plus aisément à des investissements participatifs et recevoir gratuitement des dispositifs de garantie d'origine. Tels sont, en substance, les principaux apports du Sénat

Je souhaite qu'elle contribue puissamment à inscrire le Parlement au coeur des enjeux énergétiques et climatiques. Il y va du devenir de notre modèle socio-économique, mais aussi, je le crois, de celui de nos institutions démocratiques !

le projet de loi qui nous réunit ce matin sera un texte important pour notre politique climatique et énergétique. Il constitue un nouveau pilier de nos objectifs énergétiques et climatiques. Il inscrit pour la première fois la neutralité carbone au niveau législatif. Plus important encore, il nous donne de nouveaux leviers pour atteindre ces objectifs : réduire nos émissions de gaz à effet de serre, diminuer nos consommations, développer les énergies renouvelables et lutter contre les passoires thermiques. On avait reproché à ce projet de loi sa brièveté ; les débats ont permis de l'enrichir. Je salue le travail des parlementaires pour le renforcer et le compléter. Je remercie également la commission mixte paritaire du remarquable travail qu'elle a mené, afin d'aboutir au texte qui vous est soumis ce matin, adopté par l'Assemblée nationale le 11 septembre dernier. L'engagement pour relever le défi climatique, mesdames, messieurs les sénateurs, nous le partageons. C'est bien pourquoi le Président de la République a placé l'écologie au coeur de l'acte II du quinquennat. il l'a rappelé à l'Assemblée générale des Nations unies ces derniers jours, nous devons mettre l'impératif climatique au coeur de toutes nos stratégies et politiques.

Forts de la prise de conscience de tous sur les sujets écologiques, nous devons être déterminés. Je le suis, pour trouver des réponses concrètes et réaliser les transformations nécessaires. Ces réponses, nous devons les construire collectivement, parce que la transition écologique et solidaire est l'affaire de tous. Avec ce texte, la direction est claire : atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Pour y parvenir, il nous faut dès à présent redoubler d'efforts. Il s'agit, d'abord, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles

Mais le texte ne se contente pas d'assurer l'arrêt des centrales : il nous donne les moyens d'accompagner les territoires et les salariés- chose indispensable, car la transition écologique ne sera possible que si elle est solidaire.

qui, d'une part, précise et élargit les obligations d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture et, d'autre part, permet leur installation sur les délaissés autoroutiers. La France s'engage pleinement dans le développement à grande échelle des énergies renouvelables. Ainsi, nous allons accélérer le déploiement de l'éolien en mer.

La filière industrielle a maintenant toutes les cartes en main pour démontrer que la transition écologique est bonne aussi pour les territoires et pour les emplois. La chaleur constitue également un vecteur important de diversification de notre mix énergétique. À compter de 2022, les réseaux de chaleur seront automatiquement classés, afin de systématiser le recours à ces derniers quand ils existent. Toutes ces ambitions ne se réaliseront pas sans une révision de la gouvernance et de l'évaluation de notre politique climatique. C'est pourquoi le présent texte crée le Haut Conseil pour le climat, instance d'expertise scientifique indépendante capable d'analyser l'ensemble des politiques publiques et qui pourra se prononcer sur leur conformité à nos objectifs. C'est un gage de transparence pour l'État et un outil pour nourrir le débat public. Je me réjouis également du rôle accru qu'exercera le Parlement en la matière : à partir de 2023, il établira tous les cinq ans les principaux objectifs de notre politique énergétique. Si la transition écologique est l'affaire de tous, elle est, évidemment, l'affaire de la représentation nationale. Évaluer l'impact écologique de nos politiques, c'est aussi évaluer l'incidence environnementale de nos lois de finances, en particulier leur compatibilité avec les engagements de la France- je pense singulièrement à l'accord de Paris. Le « budget vert » était un engagement pris lors du premier Conseil de défense écologique ; il est maintenant inscrit dans la loi. Il s'agit là d'une démarche inédite. Le rapport rendu hier par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable apporte une première contribution méthodologique à cette démarche, qu'il convient maintenant d'affiner. La finalité est claire : nous assurer que notre budget nous permet de respecter nos engagements, notamment l'accord de Paris.

avoir parlé d'objectifs et de gouvernance, je souhaite insister sur un élément très concret de ce texte : la lutte contre les passoires thermiques, parfaite illustration de l'ambition d'une écologie qui apporte des réponses concrètes pour améliorer le quotidien. Le logement représente plus du quart de notre consommation énergétique. Nous ne pourrons donc pas réussir la transition énergétique sans nous attaquer à la rénovation énergétique du secteur résidentiel. 4 millions de ménages modestes vivent dans des passoires thermiques et que près de 15 % des Français ont froid l'hiver dans leur logement, il s'agit d'un enjeu majeur pour la transition énergétique, mais aussi pour la qualité de vie des Français et pour leur pouvoir d'achat. Nous avons un objectif clair : la fin des passoires thermiques en 2028. Le texte prévoit un déploiement progressif des obligations de rénovation pour permettre aux propriétaires de s'adapter. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté des millions de foyers. Il nous faut accompagner les ménages, mieux les informer et leur donner confiance dans la rénovation énergétique. Les audits seront obligatoires dès 2022 pour les passoires thermiques, afin de connaître les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de ces logements. Sur ce pilier majeur de la transition, nous ne pouvons pas laisser des pratiques douteuses et de mauvaises rénovations instiller le doute chez nos concitoyens. C'est pourquoi ce texte renforce également la lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie, pour que chaque rénovation soit réellement utile pour les occupants des logements et pour le climat. mesdames, messieurs les sénateurs, depuis plusieurs mois, les marches pour le climat s'intensifient. Vendredi dernier, à Paris et dans le monde entier, notre jeunesse nous a de nouveau exhortés à agir. La mobilisation de l'ensemble de la société pour l'urgence climatique est de plus en plus visible. Comme un symbole, ce texte a été examiné à l'Assemblée nationale pendant la période de canicule de la fin du mois de juin, et la commission mixte paritaire s'est réunie alors que les températures atteignaient 45 degrés. Aujourd'hui, avec ce texte, la représentation nationale et le Gouvernement décrètent l'urgence écologique et climatique et y apportent des réponses concrètes. Pour être au rendez-vous du défi de la transition écologique, nous avons la responsabilité d'agir sur tous les leviers, du plus petit au plus grand, de l'individuel au collectif, de l'isolation thermique des logements à la fermeture des centrales à charbon. Telle est notre ambition ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre,

Car ce projet de loi entend bien, dans la continuité du plan climat présenté par le Gouvernement en 2017, concrétiser l'ambition française de la transition écologique,

Sur la forme, je salue le travail de concertation entre l'Assemblée nationale et le Sénat et me félicite que cette concertation ait permis d'aboutir à une commission mixte paritaire conclusive. l'heure où nos concitoyens attendent des réponses rapides et des engagements ambitieux, il aurait été inadmissible de se perdre dans une procédure sans fin qui, au bout du compte, aurait lassé nos concitoyens. J'espère que la mise en place d'une loi quinquennale fixant les grands objectifs de la politique énergétique

Sur le fond, le groupe Union Centriste est satisfait des avancées contenues dans ce projet de loi, qui entérine la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, développe de nouveaux outils de pilotage de la politique climatique et renforce la maîtrise du prix de l'énergie. Le rapporteur l'a très bien expliqué : ce texte replace le rôle du Parlement sur la politique stratégique en matière d'énergie et de climat, en actualisant les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2020,

Le groupe Union Centriste se félicite également des apports du Sénat à ce projet de loi, en particulier pour encourager le développement de sources d'énergie alternatives dans le mix énergétique national, qu'il s'agisse de l'hydroélectricité, du biogaz, de l'éolien ou du recours facilité à un plus grand nombre d'installations photovoltaïques. Le Sénat a aussi fait des propositions visant à encourager la montée en puissance des acteurs locaux, en facilitant les projets d'autoconsommation collective, en renforçant la cohérence entre les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid et les plans locaux d'urbanisme et en mettant en oeuvre des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. Sur cette question de la rénovation thermique des logements, permettez-moi d'exprimer une certaine déception. Car si notre gouvernement affiche l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050, cela implique à la fois d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or le secteur du bâtiment représente à lui seul 43 % de la consommation d'énergie finale en France.

De même, la question de ce que nous avons coutume d'appeler les passoires thermiques souligne la résonance entre précarité énergétique et inégalités sociales : la transition écologique peut et doit être au service des plus défavorisés, pour améliorer leurs conditions de vie et réduire les inégalités.

L'examen prochain du projet de loi de finances sera l'occasion pour le Gouvernement de manifester et de traduire dans les faits son ambition en matière d'action Plusieurs enseignements sont à tirer de ce projet de loi et, plus globalement, de la stratégie nationale bas-carbone, de la programmation pluriannuelle de l'énergie et des politiques publiques qui en découlent. Tout d'abord, le financement de ces politiques repose essentiellement sur le consommateur final, ce qui rend l'effort supplémentaire pour le financement de la transition écologique moins acceptable par nos concitoyens et explique l'impératif de pédagogie que j'ai évoqué au début de mon intervention. La remise en cause de l'augmentation de la taxe carbone en est un exemple criant. Par la suite, de telles politiques publiques devront s'accompagner d'un pendant industriel permettant l'émergence de technologies et de filières nationales stratégiques et favorisant le développement de programmes d'alliances industrielles sur le modèle de l'« Airbus des batteries Enfin, les mesures contenues dans le présent projet de loi, fortement axées sur l'offre, pourraient être complétées par un volet consacré aux économies d'énergie, puisque l'énergie la moins carbonée reste celle qui n'est pas produite la présidente, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte qui va dans la bonne direction et réaffirme l'ambition de notre politique énergétique. Mais ne nous voilons pas la face : les enjeux et défis sont si transversaux qu'il importe d'agir avec la même ambition et la même exigence dans d'autres domaines, qu'il s'agisse des mobilités, de l'économie circulaire, du verdissement de notre budget, ou encore d'une politique européenne ambitieuse dans ce domaine. À cet égard, je me réjouis que la nouvelle commission européenne ait promis la première loi européenne pour le climat, afin de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone dès 2050 ! La parole

le projet de loi que nous examinons ce matin entend répondre à l'urgence climatique par la redéfinition de la politique énergétique de la France. Nous n'avons certes pas de temps à perdre. Cependant, nous regrettons que le Sénat ait été contraint d'examiner ce projet de loi relatif à l'énergie et au climat dans un temps si restreint. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable de notre rapporteur, cher Daniel Gremillet. Malgré ces difficultés, nous nous sommes attachés à enrichir ce texte. La première lecture en a d'ailleurs considérablement augmenté le nombre d'articles. La commission mixte paritaire a réalisé un travail remarquable en parvenant à un accord qui,, n'allait pas forcément de soi. Un élément fondamental a cependant fait consensus dans les deux assemblées, il convient de s'en féliciter : l'Assemblée nationale et le Sénat ont rappelé qu'il appartient dorénavant au Parlement de déterminer la stratégie. Ce sera désormais le cas, puisqu'à partir de 2023 nous fixerons tous les cinq ans les objectifs de la politique énergétique de la France. Le projet de loi comporte des dispositions qui vont, selon nous, dans le bon sens. Parmi celles-ci, l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 nous paraît extrêmement important, de même que celui de réduction à 40 % de la part des énergies fossiles. Nous soutenons également la composition d'un bouquet énergétique provenant de différentes sources permettant d'assurer une complémentarité, mais aussi une fiabilité de l'approvisionnement énergétique. Ce bouquet doit comprendre une part croissante

et que des panneaux solaires ne puissent pas être installés sur les sites dégradés des zones littorales, nos littoraux devant être préservés. Nous croyons aussi que le développement des énergies renouvelables doit se faire au côté de l'énergie nucléaire. La France dispose en effet d'un atout majeur dans la production d'électricité décarbonée. En 2016, la production française d'électricité générait ainsi cinq fois moins de CO2 que la moyenne de l'Union européenne ; il faut savoir le rappeler. L'énergie nucléaire doit cependant être elle aussi strictement encadrée : il ne faudrait pas que le prolongement de l'exploitation des centrales se fasse au détriment de la sécurité. Enfin, le renforcement des contrôles contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie nous paraît nécessaire. Il faudra cependant veiller à assurer une visibilité et une stabilité du dispositif pour les acteurs vertueux de ce système qui fonctionne. Pour s'accorder sur une version commune, il a fallu parvenir à des compromis. Il demeure ainsi des points qui auraient pu être améliorés. Au sujet notamment des certificats d'économies d'énergie, il nous semblait légitime que le Parlement, et non l'exécutif, De même, nous aurions souhaité que la possibilité pour les parlementaires de saisir le Haut Conseil pour le climat soit conservée. Nous regrettons aussi qu'il ne soit plus prévu qu'un membre du Haut Conseil soit saisi en fonction de ses connaissances les impacts du dérèglement climatique dans les territoires ultramarins, territoires particulièrement exposés. Le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera en faveur de ce texte issu des travaux la commission mixte paritaire parce qu'il contient des mesures utiles à la protection de l'environnement.

Je me réjouis que le Sénat ait pu trouver un accord avec l'Assemblée nationale sur ce projet de loi aux enjeux cruciaux. Tout au long de nos travaux parlementaires, les débats, nombreux et constructifs, ont permis d'enrichir considérablement le texte et de prévoir les outils pour agir face aux dérèglements climatiques. Sans être exhaustive, je souhaite revenir sur les avancées majeures qu'apporte ce texte. Tout d'abord, il réaffirme et renforce nos objectifs en termes de décarbonisation de notre production énergétique, avec comme ambition la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il nous faut maintenant redoubler d'efforts, et, en premier lieu, réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Avec ce texte, l'ambition de réduction de ces énergies est non plus de 30 %, mais de 40 % d'ici 2030- les quatre dernières centrales à charbon seront fermées prochainement -, et l'accompagnement des salariés et des territoires est prévu. C'est indispensable : la transition écologique ne sera possible et acceptée que si elle est solidaire. L'atteinte de ces objectifs ne sera rendue possible également que par le développement d'énergies propres. Pour atteindre la neutralité carbone, nous devons accroître considérablement notre production d'énergies renouvelables. De manière cohérente avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce texte permet d'augmenter la production hydroélectrique, la part du solaire, ou encore les capacités de l'éolien en mer. Ces objectifs ambitieux s'inscrivent dans une stratégie globale se voulant réaliste et pragmatique. Ainsi, la date à laquelle la part du nucléaire atteindra 50 % dans la production électrique est décalée de 2025 à 2035. Au-delà de la production énergétique, c'est tout notre rapport à la consommation que nous devons changer. Notre consommation énergétique au sein du logement doit être au centre de notre préoccupation. Elle représente près de la moitié de notre consommation d'énergie nationale, et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi prévoit un dispositif d'obligation de rénovation des passoires thermiques dont le déploiement sera progressif dans le temps pour mieux permettre aux propriétaires de s'adapter. Par ailleurs, et c'est une grande victoire, c'est désormais au Parlement de fixer les priorités d'action de la politique énergétique de la France.

Chaque loi quinquennale pour la politique énergétique devra notamment prévoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz, ou encore la diversification du mix de production d'électricité. Mes chers collègues, ce texte de loi est un premier pas ambitieux et résolument tourné vers l'avenir. Il représente un nouveau pilier de notre ambition pour la transition écologique, et sera renforcé par le projet de loi d'orientation des mobilités, le projet de loi de finances et le suivi du Haut Conseil pour le climat. Grâce à ce texte, nous disposons de leviers concrets pour atteindre nos objectifs. L'engagement pour relever le défi climatique, nous le partageons tous. Forts de cette prise de conscience commune sur la nécessité d'une accélération écologique, nous devons être déterminés. Parce que la transition écologique est l'affaire de tous, ce texte ne réglera pas tout : nous devons trouver et construire collectivement avec la société civile, les territoires et les partenaires sociaux les réponses concrètes pour promouvoir les transformations nécessaires. Le groupe La République En Marche votera en faveur de l'accord trouvé sur le présent projet de loi. Tournons-nous désormais vers le projet de loi de finances qui permettra de finaliser les aspects financiers. La parole

ces faits, ce sont les incendies qui ont ravagé une immense partie de la forêt amazonienne, ressource formidable de biodiversité et de carbone vital-forêt primaire dans laquelle, en Guyane, vous autorisez toujours des exploitations minières tout en niant le droit des peuples autochtones. Autre alerte, les nouvelles simulations qui serviront de base au rapport du GIEC de 2021 prévoient que la hausse de température moyenne globale pourrait atteindre 6,5 à 7 degrés en 2100. Pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés en 2040, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre devraient être immédiates et massives, sans commune mesure avec les trajectoires actuelles, ni même avec les engagements- non respectés d'ailleurs -de l'accord de Paris. L'objectif de 40 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 est donc bien insuffisant pour rester sous 2 degrés de réchauffement et atteindre une neutralité carbone en 2050. Les scientifiques nous ont alertés de nouveau hier lors de la présentation du rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur nos océans. Elles sont catastrophiques amoindrissement des capacités d'absorption du CO2 par l'océan, disparition des écosystèmes marins, hausse du niveau des mers ... Le changement climatique n'est plus une menace théorique il est déjà une réalité. Si rien n'est fait, à terme, et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, toutes les espèces, la nôtre incluse, seront menacées. Madame la ministre, nous n'avons plus confiance. Les jeunes, les ONG, les gilets rouges, jaunes ou verts n'ont plus confiance non plus. Ils ont compris une chose vous ne changez rien et vous ne changerez rien. Vos mots sonnent creux et marquent votre impuissance. Vos politiques restent soumises au capitalisme, à la surconsommation à outrance et à la course au profit. Pourtant, agir n'est plus une option : c'est un impératif vital, qui implique des changements radicaux, globaux et rapides. En premier lieu, il est nécessaire de rompre avec l'austérité budgétaire pour investir largement. Ainsi, une stratégie globale de lutte contre le changement climatique ne peut se limiter à la production d'électricité, mais doit porter également sur l'efficacité énergétique, le logement, les transports, l'alimentation, bref tous les étages. Il est facile de se donner bonne conscience en déclarant l'urgence climatique à l'ONU ou de faire des selfies tout l'été avec le cacique Raoni. Mais où sont les milliards d'euros nécessaires à la transition énergétique ? Assurément pas dans ce projet de loi Où sont les filières industrielles pour la réussite de la transition énergétique ? Assurément pas en France ! Le Haut Conseil pour le climat fait état d'un manque d'investissements publics et privés de plus de 40 milliards d'euros en 2018 dans les secteurs clés des transports, du bâtiment et de la production d'énergie. En parallèle, les investissements qui entretiennent l'utilisation des énergies fossiles en France ont atteint 75 milliards d'euros en 2017 ! C'est sûrement la politique du « en même temps Il est nécessaire également de rompre avec le libre-échange et la multiplication d'accords commerciaux accroissant consumérisme, transport international de marchandises et dumping environnemental. Madame la ministre, vous voulez sauver l'Amazonie et la planète ? Alors ne signez pas le Mercosur et le CETA qui vont accélérer l'agro-business et la déforestation ! L'astrophysicien Jean-Pierre Bibring rappelait lors de la dernière Fête de l'Humanité que « nous consommons sur terre plus d'énergie qu'en produit le noyau terrestre. Sans changement de mode de production, de consommation, sans la fin du capitalisme tel que nous le connaissons, ce sera la fin de nos civilisations. Il nous faut sortir du " capitalocène Ces menaces pesant sur la planète creusent également les inégalités entre continents, entre pays et dans chacun d'entre eux. La précarité s'installe durablement en France, et avec la fin des tarifs réglementés du gaz et la prise en compte de l'atteinte du plafond de l'Arenh dans le calcul des tarifs réglementés de vente d'électricité, elle sera accentuée. Ce texte maintiendra de nombreuses familles dans des passoires thermiques tant les reculs sur le volet logement ont été importants. Voici la réalité : ce sont les plus précaires qui subissent en premier lieu le réchauffement climatique. Ce qui anime ce projet de loi, c'est la poursuite du démantèlement général du service public, de l'énergie, à travers la promotion des communautés d'énergie et la fin des tarifs réglementés. Or la transition énergétique ne se fera pas sans justice sociale. Pour conclure, la lutte contre le changement climatique ne peut être de la seule responsabilité des individus. Il faut un engagement massif des États et des entreprises. Ce projet de loi aurait dû être l'occasion de prendre la mesure de l'urgence à laquelle nous sommes tous confrontés. Je citerai pour finir Philippe Geluck, le père de la bande dessinée : « Je pense sincèrement que la pollution de la planète, ce n'est pas aussi grave qu'on le dit

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je l'ai déjà dit, ce qui se joue désormais au niveau planétaire, c'est la survie de l'humanité. Avec une hausse possible de 7 degrés en 2100 selon les scénarios les plus pessimistes, le pire est de plus en plus sombre. Tout va donc dépendre des politiques qui seront mises en oeuvre dès maintenant à l'échelon de la planète. L'objectif de maintenir l'élévation de la température à 2 degrés ne relève pas de la pure convenance. Il est temps que le climat soit perçu comme un enjeu d'intérêt général majeur et de survie. Il s'agit non pas d'en rajouter dans le registre anxiogène, mais de nous mobiliser, sans oublier que transition énergétique et justice sociale doivent être étroitement liées. Pour la première fois dans l'histoire, l'histoire, détruit les conditions mêmes de sa vie sur Terre. La France n'est pas forcément le plus mauvais élève, mais reconnaissons que nous pourrions faire bien mieux. Avec ce texte, peut-on dire que notre pays se situe bien dans les clous des derniers rapports du GIEC et des scénarios les plus alarmants ? Je ne le crois pas. Ne pouvait-on attendre plus et mieux d'un tel projet reconnais toutefois qu'il permet certaines avancées et que le Sénat, monsieur le rapporteur, a été à l'origine de plusieurs d'entre elles. Il n'empêche qu'à l'issue de la CMP la régression qui en résulte, ce texte restera pour le groupe socialiste celui des occasions manquées. Pourtant, mon groupe a été animé en première lecture pas une réelle volonté de coconstruction législative. Peine perdue ! La CMP a ruiné tous nos efforts. Angèle Préville nous en dira peut-être plus sur cette entreprise de démolition. Autre question : le projet de loi prévoit-il un plan d'envergure, et surtout rapide, en faveur du sujet central qu'est la rénovation thermique des logements passoires ? Disons que cela ne nous a pas sauté aux yeux. L'urgence climatique va devoir attendre d'hypothétiques financements qui soient vraiment à la hauteur. Nous attendons donc avec impatience le prochain projet de loi de finances, madame la ministre, car avec la

une fois ! C'est dommage, car c'était pourtant une belle occasion d'apporter un cinglant démenti à ceux qui reprochent à la France de donner volontiers des leçons mais pas assez d'exemples. Je n'en rajoute pas sur la regrettable suppression ou les restrictions apportées au tarif réglementé de l'énergie, ni sur le mal que je pense de l'Arenh, mécanisme visant à créer une concurrence en réalité fausse, organisée sur le dos d'EDF, à qui on impose aujourd'hui de biberonner des concurrents comme Total, lesquels d'ailleurs se prévalent d'avoir zéro dette alors qu'EDF est déjà endetté et doit faire face à un mur d'investissements. Ne devrait-on pas parler de spoliation ? Depuis 2012, EDF a perdu 3 millions de clients. Ne doit-on pas considérer que le marché est déjà bien ouvert ? Pourquoi donc ce déplafonnement qui ne semble dès lors répondre à aucun motif d'intérêt général ? Par ailleurs, il est regrettable que la CMP ait supprimé la révision concomitante du plafond et du prix de l'Arenh proposée par le rapporteur au Sénat. Madame la ministre, y aura-t-il au moins concomitance entre le déplafonnement et la maigre prise en compte de l'inflation qui subsiste ? Enfin, nous aurons je pense l'occasion de revenir sur le projet de scission d'EDF, baptisé Hercule, véritable projet de découpe et de privatisation partielle. Pour conclure, alors que nous nous étions abstenus en première lecture, le texte issu des travaux de la CMP est tel qu'il nous conduit à voter contre,

si ensuite les politiques publiques ne sont pas mises en cohérence. Or tel a été le cas après l'adoption de la loi susvisée en 2015 : les politiques publiques n'ont pas suivi, notamment sur le développement des énergies renouvelables. La France est sur ce point, nous le savons et il faut le rappeler, largement en retard par rapport à ses engagements européens.

Avec l'abandon d'Astrid en rase campagne, ce risque paraît s'éloigner. L'EPR continue d'accumuler les déboires et semble techniquement comme économiquement totalement incapable d'incarner sérieusement un quelconque avenir pour la filière nucléaire. Il faut donc nous donner maintenant rendez-vous dans cinq ans pour la prochaine discussion de cette nature. Nous serons alors dans l'extinction progressive de cette parenthèse nucléaire. Les choses évoluent par conséquent dans le bon sens.

de l'article 6 relatif à la possibilité pour les organismes d'HLM d'organiser des projets d'autoconsommation. C'est une évolution importante. Nous soulignons aussi que l'Assemblée nationale a accepté, dans la dernière ligne droite de la CMP, de mentionner que le

c'est dans sa nature-entre vote pour et abstention, mais j'espère que vous entendrez l'abstention des sénateurs écologistes comme un signal bienveillant quant à la nécessité d'un travail en commun dans la durée, tant l'urgence climatique, je le dis très sincèrement, ne nous laisse pas le temps des postures, des phrases définitives non suivies d'effets, mais appelle à des solutions partagées ambitieuses et discutées collectivement. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à saluer le travail important qui a été accompli, malgré les délais très contraints dont nous disposions pour enrichir ce projet de loi et trouver un accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire. Par rapport à sa version initiale qui comportait huit articles et qui, il faut le rappeler, avait assez peu d'ambition, le texte de compromis qui nous est présenté aujourd'hui a été substantiellement enrichi sur de nombreux points. En tant que rapporteure pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en première lecture, je tiens à remercier le rapporteur au fond, M. Daniel Gremillet, des échanges que nous avons eus sur ce rapport. J'associe à ces remerciements les administrateurs des deux commissions. Je tiens Je tiens à le dire, je suis particulièrement satisfaite des accords que nous avons trouvés sur les articles qui avaient été délégués au fond à notre commission. Je pense notamment à l'article relatif au Haut Conseil pour le climat, dont les missions ont été confortées et précisées, et auquel nous avons donné la souplesse nécessaire pour organiser son travail, notamment, comme vous l'avez dit, madame la ministre, quant à la conformité des futurs budgets avec les objectifs environnementaux.

La volonté de confier au préfet la compétence d'examiner au cas par cas si les projets d'aménagement doivent ou non faire l'objet d'une étude d'impact environnemental laissait craindre une multiplication des recours pour conflit d'intérêts, ce qui aurait fortement insécurisé les porteurs de projets. Je suis donc satisfaite que la rédaction de compromis trouvée fasse clairement figurer dans la loi la nécessité que les autorités compétentes pour réaliser cet examen au cas par cas ne soient pas en situation de conflit d'intérêts par rapport à l'autorité chargée de valider ces mêmes projets.

cette solution qui n'était pas pertinente, car elle aurait affaibli le droit au recours, alors même qu'il existe déjà une procédure dérogatoire au droit commun. S'agissant des articles sur lesquels la commission de l'aménagement du je me réjouis que les dispositions intégrées par le Sénat pour améliorer l'accompagnement des salariés dont l'emploi serait supprimé à la suite de la fermeture des centrales à charbon et des centrales nucléaires aient été conservées.

visant à annexer à la programmation pluriannuelle de l'énergie une feuille de route relative au démantèlement des réacteurs nucléaires n'aient pas été conservées dans le texte final. Il est pourtant essentiel que l'État travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière à l'élaboration d'une stratégie de démantèlement, afin, notamment, de s'assurer du maintien de compétences techniques dans ce domaine.

Le vote d'une loi de programmation quinquennale était plus que nécessaire et permettra à nos deux assemblées de faire entendre la voix des citoyens et des territoires. Le Parlement retrouve en outre une place importante dans sa fonction de contrôle du Gouvernement, désormais une évaluation des incidences de nos lois de finances sur le réchauffement climatique. Verdir nos politiques est un enjeu majeur. Mais verdir, ce n'est pas vernir,

Le prochain débat budgétaire sera d'ailleurs l'occasion pour le Gouvernement de démontrer toute sa détermination sur le sujet. Je pense également à des secteurs énergétiques abordés à la faveur de la discussion et sur lesquels nous devons aller plus loin, comme la petite hydroélectricité et, surtout, l'hydrogène. Je pense enfin au renforcement du dispositif des certificats d'économies d'énergie, qui doit désormais entrer dans sa phase de maturité. Pour avoir moi-même appliqué ce projet en Meurthe-et-Moselle, j'en mesure toute l'importance et la portée. Le texte que nous nous apprêtons à voter après plusieurs mois de procédure législative ne règle pas tout, tant s'en faut. Pour autant, je crois que le Parlement a tenu son rôle, et nous devons collectivement nous en satisfaire. Madame la ministre, le vrai rendez-vous est pour bientôt

Je crois à une écologie pragmatique, consentie, pour laquelle des moyens sont accordés par les États. Eh oui ! C'est la raison pour laquelle, sur le soutien aux énergies renouvelables, sur la prime à la conversion, sur le chèque énergie ou sur la transformation du crédit

ce projet de loi qui devait marquer une étape majeure dans notre transition énergétique et écologique n'est ni à la hauteur des enjeux ni pourvu d'une vision globale à long terme. Je m'attacherai à vous le démontrer. Pour ce qui il s'agit principalement de la diminution des gaz à effet de serre. Je tiens à rappeler, à toutes fins utiles, que la quasi-totalité de la production électrique dans notre pays est décarbonée et n'émet donc que peu de gaz à effet de serre. Autrement dit, la fermeture des centrales à charbon, qui produisent une électricité très marginale, est un épiphénomène. En réaction à l'adoption de cette mesure,

actionné dans le texte, car les mesures sont trop peu contraignantes dans l'immédiat. Et pourtant, je vous rappelle qu'il y a urgence ! Deuxièmement, le Gouvernement doit assumer les responsabilités sociales de ses décisions. La question qui se pose aujourd'hui pour les centrales à charbon se posera par la suite pour les centrales nucléaires. Les plans de réemploi doivent être au coeur des préoccupations gouvernementales. L'époque et le contexte ambiant vous le prouvent de mille manières : le volet social doit être inclus dans les mesures d'urgence climatique. la vision maintenant, nous ne retrouvons aujourd'hui ni projet partagé ni ligne conductrice. Pourtant, le réchauffement climatique est plus rapide que prévu et l'extinction des espèces s'accélère. Les chiffres sont toujours plus alarmants et les politiques publiques insuffisamment réactives. Certes, le développement des énergies renouvelables se poursuit, mais à une vitesse trop faible et de façon trop aléatoire, voire chaotique sur le territoire. L'hydroélectricité, elle, est capable de maintenir le réseau et les fréquences. Malgré les avancées obtenues grâce au rapporteur, nous déplorons un manque d'engagement chiffré

d'abord à la suppression de la mesure relative au financement participatif des réseaux de chaleur. Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux et prévoit de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid de récupération d'ici à 2030, ce financement était un outil pertinent de développement des réseaux. à la suppression d'une possible stratégie pour le développement des projets d'énergie renouvelable détenus par les citoyens et les collectivités territoriales qui aurait été annexée à la PPE.

ouvert et fluctue. EDF continuera à perdre des parts de marché, en moyenne 100 000 clients par mois. Or le nucléaire historique tend à baisser : multiplication des arrêts du fait de centrales vieillissantes, travaux de grand carénage, sécheresse. EDF est fragilisée, car elle supporte seule les engagements et la responsabilité à long terme du nucléaire. Gardons en mémoire le risque d'accident. Notre inquiétude naît de ce que l'intérêt stratégique doit être au centre de la résolution de cette difficile équation et du futur d'EDF.

le projet de loi de finances pour 2020 traduira bien la montée en puissance des dispositifs d'accompagnement de nos concitoyens dans la transition écologique, qu'il s'agisse du chèque énergie, de la prime à la conversion, du forfait mobilité, qui sera mis en place l'an prochain, ou encore de la rénovation thermique thermique des logements. J'ai entendu vos préoccupations et votre souhait d'une politique ambitieuse dans ce domaine. Je peux vous dire que je la partage : c'est le sens des simplifications que nous sommes en train de mettre en oeuvre en matière de rénovation énergétique des logements avec un dispositif

en outre tendre vers une transformation de nos modèles de consommation. C'est le sens du projet de loi que vous examinez en ce moment même sur l'économie circulaire. Là encore, je pense que nos concitoyens sont prêts à changer leurs comportements ; ce projet de loi vise à les accompagner. faut enfin un changement de nos modèles d'aménagement pour lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Ce sont toutes ces transformations qu'il nous faudra conduire.

l'année, avec la transformation de la Banque européenne d'investissement en une Banque du climat, le verdissement du budget, dont 40 % des crédits doivent être consacrés à la transition écologique, la mise en place d'un prix du carbone à l'échelle européenne,

Or l'effacement possible est loin d'avoir mobilisé les capacités disponibles. Ne parlons même pas des critères environnementaux, qui sont fixés aux articles 6 et 62 et qui découlent des directives européennes, car ils ne sont même pas mis en oeuvre. Nous savons que cette insuffisante mobilisation de

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse

Ce texte qui réforme en profondeur l'historique loi Bichet de 1947 était attendu- c'est le moins que l'on puisse dire -et depuis longtemps, tant les principaux rouages qui ont fait la force et l'efficacité de notre système de distribution depuis la Libération étaient grippés, voire défaillants. Il vous est revenu, monsieur le ministre, de mener à bien ce chantier avec courage et, je dois le dire, avec habileté. Il y avait un point d'équilibre à trouver entre les diffuseurs de presse, trop souvent oubliés du système, les éditeurs, les deux messageries, mais également les dépositaires centraux. Sans aller jusqu'à tenter de faire croire que le texte que nous examinons aujourd'hui a satisfait tout le monde, je crois pouvoir dire qu'il constitue une position raisonnablement satisfaisante, qui offre enfin des perspectives de développement et conforte le modèle économique de la presse. Pour parvenir à cet équilibre, monsieur le ministre, vous avez choisi de vous appuyer sur le Parlement, singulièrement sur le Sénat, que vous avez saisi en premier lieu. Je tiens à souligner et à saluer votre capacité d'écoute et celle de vos services, qui, sous votre impulsion, nous ont permis de travailler en toute confiance et en toute clarté. Je n'oublie pas non plus les collaborateurs de la commission de la culture du Sénat. Je tiens à rappeler les grands principes de ce texte. Premier principe, la régulation sera intégralement confiée à l'Autorité de régulation des La nouvelle autorité de régulation devrait notamment veiller à ce que les nouvelles sociétés agréées qui assureront, à compter de 2023, la distribution des journaux sur le territoire oeuvreront bien dans le respect des objectifs d'intérêt général attachés à la presse. Deuxième principe, les diffuseurs de presse seront enfin placés au centre du système, avec la possibilité de mener une réelle politique commerciale. À l'accès illimité au réseau, ayant contribué à l'engorgement des linéaires, va succéder, une fois précisée que la presse d'information politique et générale conserve un droit absolu à être distribuée, une négociation pour déterminer l'assortiment servi dans les différents points de vente.

Cette conviction, soutenue à l'échelon européen de manière forte par notre présidente, Catherine Morin-Desailly, qui a fait adopter à l'unanimité une résolution européenne sur la responsabilité des hébergeurs, sera prochainement réaffirmée en séance avec la proposition de loi visant à lutter contre les

l'initiative de Jean-Pierre Leleux, le droit de « première présentation » des éditeurs auprès des distributeurs de presse, ce qui garantit l'accès au réseau pour toutes les nouveautés l'initiative de David Assouline, la mention dans le cahier des charges des futures messageries du respect des principes d'indépendance, de pluralisme, de non-discrimination et de continuité territoriale, ainsi que la publicité des barèmes établis par les sociétés agréées l'initiative de Françoise Laborde, la mission de veiller au respect du pluralisme confiée à l'Arcep. Monsieur le ministre, vous vous étiez par ailleurs engagé à répondre à la préoccupation exprimée par Françoise Laborde, qui souhaitait inscrire dans la loi que l'Arcep disposait heures pour répondre à une situation mettant en jeu la distribution des quotidiens. L'Assemblée nationale a donc adopté un délai de quarante-huit heures dans ce cas précis, contre un mois pour les autres publications. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir su répondre à cette préoccupation légitime et d'avoir ainsi tenu votre engagement. De son côté, l'Assemblée nationale a mené un important travail de coordination de l'ensemble des dispositions du texte. Elle a également pu traiter la question du statut des porteurs de presse, par souci d'équité avec les vendeurs colporteurs. seules deux divergences sont apparues entre nos assemblées La première concerne la problématique des dépositaires centraux. L'Assemblée nationale est revenue au texte initial, ce qui ne me paraissait pas suffisant compte tenu de la place centrale de la profession.

conforme. L'Assemblée nationale a jugé bon de revenir à un avis simple ; à la réflexion, cela me semble plus prudent. Dès lors, rien ne s'opposait à l'accord que nous avons élaboré avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, Laurent Garcia, que je tiens à saluer pour la qualité de son écoute.

Tout d'abord, à très court terme, il faudra trouver une solution à la situation de Presstalis. On parle d'adossement, mais ce dossier ne semble pas progresser. En dépit des efforts certains de l'ensemble des personnels, les comptes sont encore déficitaires. Nous avons appris très récemment le départ de la présidente de l'entreprise, Michèle Benbunan, avec laquelle nous avions travaillé en toute confiance. L'examen du prochain projet de loi de finances pourra nous offrir l'occasion de dresser un état de la situation, mais je constate, à regret, qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis le mois d'avril. Or la distribution de quotidiens repose aujourd'hui sur cette seule société et il serait illusoire de penser que son défaut aurait une incidence autre que désastreuse pour toute la filière. À moyen terme, il faudra répondre aux défis posés par l'adaptation du réseau des vendeurs de presse. Ces derniers ont été trop longtemps les grands oubliés d'un système plus axé sur la distribution que sur la vente. L'amélioration de leurs conditions d'exercice et de leur niveau de vie doit rapidement découler de la mise en place du nouveau système issu du texte que nous examinons ce jour. Il faudra, pour ce faire, que les éditeurs et les messageries jouent rapidement le jeu, mettent à niveau un système informatique très défaillant et soient en mesure de nouer un dialogue commercial suivi et fluide. J'en profite pour dire un mot sur le rôle, qui me paraît essentiel en la matière, des dépositaires centraux de presse. Ceux-ci constituent un maillon indispensable à ce jour, et je suis heureux de pouvoir dire que le compromis trouvé avec l'Assemblée nationale s'est traduit par un geste en leur faveur. Enfin, à plus long terme, il faudra s'assurer que les principes mis en place d'ici au 1 janvier 2023, et désormais soumis au contrôle de l'Arcep, puissent pleinement s'appliquer au bénéfice de tous et qu'ils permettront de mettre un terme, comme je le souligne depuis longtemps, aux renflouements réguliers

partagé par tous. En conclusion, si le secteur de la presse traverse une crise, dont nous avons tous conscience, nous avons su collectivement, et avec un grand sens des responsabilités, nous emparer de ces sujets et commencer à les traiter avec enthousiasme et dans des délais très brefs. Nos débats ont souvent montré de réelles convergences, traduisant bien l'attention que nous portons à la liberté et à l'indépendance de la presse. ici, la proposition de loi de notre collègue David Assouline tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, adoptée à l'unanimité par le Sénat et adoptée conforme par l'Assemblée nationale. Ce texte offre de réelles perspectives, dont doivent maintenant se saisir les acteurs de la presse.

mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous y voilà ! J'entends encore ceux qui disaient la réforme de la loi Bichet impossible à mener ... Pourtant, nous l'avons fait ! Vous l'avez fait

; de votre souci constant de clarifier, de préciser, de rendre plus lisible le texte du projet de loi initial. Vous l'avez sensiblement amélioré, et vous l'avez fait dans le consensus, avec un esprit résolument constructif. Merci à tous, infiniment

Face aux difficultés économiques rencontrées par la presse- notamment Presstalis -, il devenait indispensable de moderniser sa distribution. Mais il fallait la moderniser, tout en prenant soin de ne pas casser les acquis du système actuel. évidemment pas été tâche aisée. Je crois néanmoins que le projet de loi présenté par le Gouvernement parvient à résoudre cette équation. Il permet de préserver les grands principes de la loi Bichet : le principe coopératif obligatoire, le droit absolu à la distribution de l'ensemble des titres d'information politique et générale et donc,, l'accès pour nos concitoyens à une diversité de publications sur l'ensemble du territoire. Cette diversité est garante du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Elle est une condition d'effectivité de la liberté de la presse. Le dernier rapport de Reporters sans frontières, publié hier, le rappelle avec force : attenter à la distribution de la presse est une méthode tristement classique pour attenter à la liberté de la presse elle-même. Je le disais, le projet de loi préserve ces principes. Mais, dans le même temps, il propose une vraie modernisation du cadre législatif. Il met en place un nouveau cadre de régulation, indépendant, cohérent et renforcé. Il donne aux marchands de journaux une plus grande marge de manoeuvre dans le choix des titres qu'ils distribuent, en dehors, bien sûr, de la presse d'information politique et générale et des assortiments de la presse reconnue par la Commission paritaire des

Enfin, il garantit la continuité de la distribution de la presse, en laissant aux deux principales messageries aujourd'hui en service un temps d'adaptation suffisant avant l'arrivée éventuelle de nouvelles sociétés de distribution. la possibilité pour l'Arcep, futur régulateur, de délivrer des agréments à d'autres acteurs que les deux opérateurs actuels ne pourra intervenir qu'après une phase de transition.

Merci à vous tous pour votre engagement ! La commission mixte paritaire de mardi a été conclusive. Je me réjouis, au nom du Gouvernement, de l'obtention de cet accord, ouvrant la voie à une promulgation rapide de la loi. Conformément à l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement soumet donc à votre approbation le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'avenir de la presse dépend en grande partie Mais il dépend également d'un juste partage de la valeur créée, de la juste rémunération des éditeurs et agences de presse par les plateformes, lorsqu'elles réutilisent leurs contenus. C'est l'objet de la loi tendant à créer un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse.

travail au service de la presse et de l'information de nos compatriotes. Je m'entretiendrai par conséquent prochainement avec mes homologues européens pour remédier à cette situation. Vous l'avez souvent rappelé, chère Catherine Morin-Desailly, cher David Assouline, nous devons travailler à une refonte de la directive e-commerce pour une véritable responsabilisation des plateformes.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie mardi 24 septembre dernier, est parvenue à un accord, sans surprise tant la réforme de la loi Bichet est attendue. C'est le signe que nos assemblées peuvent se retrouver sur des positions communes et travailler de façon constructive avec le Gouvernement, pour sauver- ou défendre, plutôt -un des symboles de notre démocratie : la liberté de la presse. présent texte est décisif pour la survie d'un secteur en crise, qui doit maintenant se moderniser pour franchir le cap de la révolution numérique. La chute du volume de vente au numéro de 54 % en dix ans, l'attrition des revenus de la presse écrite de 41 % sur la même période, la fermeture des points de vente, au rythme de 1 000 par an, sont les principaux symptômes de cette crise ayant touché de plein fouet la principale messagerie de presse, Presstalis. En réponse à cette situation d'urgence, le Gouvernement a fait le choix d'ouvrir le secteur de la distribution à la concurrence à l'échéance de janvier 2023 et de placer la régulation du secteur sous la responsabilité unique de l'Arcep, dont les pouvoirs, renforcés, seront étendus aux kiosques numériques. Pour offrir plus de souplesse aux marchands de presse dans la gestion de leur commerce, le Gouvernement a aussi fait le choix d'instaurer une quasi-liberté d'assortiment des titres. Cette liberté n'est pas absolue. D'une part, le texte institue un principe de non-discrimination et de transparence au profit de la distribution des publications. D'autre part, l'accès des éditeurs de titres d'information politique et générale à l'ensemble du réseau de distribution est une garantie constitutionnelle qu'il n'est pas question de remettre en cause. Il s'agit de préserver le pluralisme des opinions et la vitalité des débats, et nous en mesurons l'importance. Ainsi, le Gouvernement a opté pour une évolution de la loi Bichet, sans rupture avec les grands principes qui ont sous-tendu son adoption, à l'heure de la libération de la France, comme des garde-fous démocratiques contre le déchaînement de la propagande. Ces principes sont plus que jamais d'actualité. Pour reprendre les mots du Conseil national de la Résistance, il nous faut veiller à garder intacts « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances de l'argent et des influences étrangères ». À ce titre, mon groupe se félicite de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement républicain visant à restreindre les parts pouvant être détenues par un actionnaire extracommunautaire dans une société de distribution de presse. Cette disposition vise précisément à limiter l'immixtion de puissances étrangères, États ou multinationales, dans ce que notre démocratie a de plus sensible : l'opinion publique. en effet, est une proie facile pour les algorithmes des géants du web, les Gafam, créateurs de bulles informationnelles dans lesquelles seules les opinions semblables se rencontrent et se cristallisent.

au vote de ce jour -a souhaité associer le maire à la décision d'implantation sur sa commune d'un diffuseur de presse, placée sous la responsabilité de la Commission du réseau. Le Sénat a également renforcé les pouvoirs de l'Arcep, afin de favoriser l'efficacité de la régulation du secteur et sa transparence, notamment à l'égard du Parlement et des organisations professionnelles des diffuseurs de presse, qui seront consultées avant de fixer le cadre de leur rémunération. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte va dans le bon sens. Nous savons que l'avenir de la distribution de la presse dépend de son adoption. Nous ne pouvons que le souligner et soutenir cette réforme. La parole

La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. [ ...] Pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente

Préserver une diffusion libre et impartiale de la presse écrite sur l'ensemble du territoire national représente un facteur essentiel de ce pluralisme et de la diversité À cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter de l'accord trouvé entre nos deux assemblées sur ce projet de loi, qui a fait l'objet de simples modifications quasi rédactionnelles. Saisi en première lecture, le Sénat s'est efforcé d'apporter des améliorations, que je crois notables. Je me permettrai d'en rappeler quelques-unes. D'abord, nous saluons la possibilité, prévue par le Sénat, que certains titres fassent l'objet d'une première proposition de distribution auprès auprès des points de vente. Derrière l'apparente technicité de cette disposition, se cache en réalité un objectif simple, mais essentiel : mettre les diffuseurs de presse en situation de pouvoir choisir, en parfaite connaissance de cause, les titres qui viendront compléter leur offre de presse, en plus des titres à la diffusion desquels ils ne peuvent s'opposer. Cette possibilité profitera tant aux diffuseurs de presse, leur permettant de s'affranchir des contraintes antérieures- ils revendiquaient d'ailleurs cela depuis longtemps qu'aux consommateurs, qui se verront proposer une offre mieux adaptée à leurs attentes. Par ailleurs, le Sénat a prévu que le Parlement puisse saisir l'Arcep pour avis sur toute question relative au secteur de la presse. Il semble particulièrement opportun que les commissions parlementaires concernées, développent une certaine compétence au fil de leurs travaux, puissent l'enrichir de l'expertise de l'Arcep, notamment lorsqu'elles étudient des textes de loi concernant la distribution de la Si nous ne pouvons que nous réjouir de ce que le texte du Sénat a été accueilli par les députés comme un texte « équilibré », ayant fait l'objet d'un « examen minutieux et constructif », il faut également saluer les améliorations apportées par l'Assemblée nationale. Ainsi, et à titre d'exemple, les députés ont limité à 20 % le nombre de parts pouvant être détenues par un actionnaire extracommunautaire dans une société de distribution de presse, dans le but de se garantir contre une influence étrangère trop importante. La presse constitue effectivement un atout stratégique pour notre pays et représente, de surcroît, un enjeu démocratique majeur. Cependant, bien que ce projet de loi nous semble constituer une réponse pragmatique à la crise que traverse la distribution de la presse, un impératif et des difficultés demeurent. L'impératif, qu'il nous faudra surveiller de près, c'est la mise en oeuvre effective de la future loi. Sans cela, la modernisation de la loi Bichet restera lettre morte ! Les difficultés, quant à elles, ont trait à Presstalis- son cas a été évoqué et nous sommes tous conscients de ces aujourd'hui encore, reste proche de la faillite et le présent projet de loi ne traite pas de sa situation financière. Pour cette raison, je m'interroge sur les options envisagées par le Gouvernement en vue de redresser la société. « La libre communication des pensées et des opinions est », indique la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en son article 11, « un des droits les plus précieux de l'Homme ». à protéger ce précieux droit ! Bien évidemment, mon groupe se réjouit du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera ce projet de loi, fruit d'un travail parlementaire mené en bonne intelligence, tout particulièrement

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d'une procédure parlementaire menée avec le sentiment d'une certaine urgence. Le secteur de la presse connaît de profondes mutations, comme l'ont rappelé de nombreux orateurs, mais ce texte est malheureusement loin d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Le développement du numérique a bouleversé l'économie du secteur, en participant à l'effondrement des ventes de la presse papier et, en toute logique, à l'explosion des invendus dans les kiosques. Il en va de même de l'arrivée sur le marché de l'information des Gafam, qui, sous couvert d'un statut intermédiaire de mise en relation, subtilisent le travail de la presse traditionnelle. Certes, quelques avancées pour lutter contre les effets les plus néfastes de ces bouleversements, comme la mise en place d'un droit voisin, doivent être saluées. Mais Google, cela vient d'être souligné, a annoncé hier n'avoir aucune intention de se conformer à l'esprit de cette loi, préférant la contourner allégrement. De telles réactions rappellent qu'il nous appartient de légiférer courageusement pour faire respecter la souveraineté démocratique.

mais, précisément, il faudrait adapter une législation dont les fondements ont été établis au moment de la Libération, et non rompre avec les valeurs défendues à l'époque, qui ont permis de développer notre système de distribution. le système défini par la loi Bichet garantit la liberté d'accès au réseau de distribution, l'égalité et la solidarité entre les coopérateurs. Il est synonyme d'égalité d'accès à l'information sur tout le territoire, de démocratie et de pluralisme. Ces enjeux sont bien trop déterminants dans la vie d'une démocratie pour que la presse soit traitée comme une vulgaire marchandise : c'est ce que traduit l'esprit de cette loi fondatrice, et nous serions bien inspirés de ne jamais le perdre de vue.

À ce titre, je ne peux m'empêcher de souligner que les effets délétères de la libéralisation ne tarderont pas à se manifester, à commencer par le dépérissement de Presstalis,

Le pluralisme, grande avancée du système Bichet, est lui aussi menacé par ce texte. La structure pyramidale qui va être mise en place pourrait conduire à ériger des barrières tarifaires pour les petits titres ou ceux qui sont jugés peu rentables, en opposition au système universel et solidaire actuel. on peut se féliciter que l'Assemblée nationale ait adopté le principe en vertu duquel l'Arcep s'appuiera sur les acteurs du secteur, comme nous le demandions. Mais nous restons circonspects quant à la nouvelle place accordée à cette agence. Non seulement vous écartez les principaux acteurs de la gouvernance du secteur, mais vous placez de fait la régulation de la distribution de la presse sous le signe du respect de la concurrence libre et prétendument non faussée, plutôt que de considérer l'information comme un enjeu majeur du fonctionnement démocratique. de ce renversement symbolique, on peut douter que cette nouvelle gouvernance soit réellement plus efficace que la cohabitation entre le Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse,

Loin d'adapter les principes fondateurs de la distribution de la presse aux enjeux du XXI siècle, il n'accompagne pas davantage la presse écrite dans les bouleversements qu'elle subit. Au contraire, il ouvre la voie à une inégalité territoriale renforcée et à un affaiblissement du pluralisme, qui sera lourd de conséquences sur la vie démocratique. La crise de confiance que traverse notre société rend pourtant indispensables les efforts pour une diffusion plurielle et large de l'information. Ce texte est un rendez-vous manqué,

à aimer nous référer à notre riche histoire parlementaire, où l'on puise parfois de belles leçons sur la fabrication de la loi. C'est le cas pour la loi Bichet, qui après des débats très animés sur les modalités du démantèlement du monopole d'Hachette a jeté, dès 1947,

qu'il en soit, il a suivi l'esprit du programme du Conseil national de la Résistance, et nous saluons le choix du Gouvernement d'avoir maintenu ce cadre législatif. Monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé : en 1947, il s'agissait principalement de garantir une distribution indépendante de la presse, afin qu'elle ne puisse dépendre de nouveau du bon vouloir d'un opérateur à la merci du pouvoir politique. La réponse du législateur de l'époque avait été particulièrement innovante, puisqu'elle établissait un système coopératif unique au monde. La question qui nous est posée aujourd'hui est légèrement différente : il convient d'adapter économiquement ce système aux évolutions technologiques et à la diversification des modes d'information de nos concitoyens. l'émergence de la télévision et d'internet a durablement affecté les ventes de titres de presse nationaux, la presse régionale réussissant à tirer son épingle du jeu. Notre presse d'information politique et générale a, semble-t-il, tardé à adapter son modèle économique à la diffusion en ligne, par rapport aux grands titres de la presse anglo-saxonne. En outre, les dysfonctionnements liés à la situation monopolistique de Presstalis ont aggravé le décalage entre le mode de vie des Français, qui l'immédiateté tient désormais une place importante, et la livraison de titres papiers, parfois perçue comme archaïque. Ces dysfonctionnements ne sont d'ailleurs pas sans conséquences économiques pour les points de vente qui quadrillent nos territoires. donc avec satisfaction que ce texte met un terme à quelques anomalies, en particulier le maintien d'un acteur économique défaillant comme Presstalis l'est devenu. S'il avait été confronté à la seule loi du marché, il n'existerait probablement plus aujourd'hui. Ce projet de loi permet également de prévenir les dévoiements constatés du fait de l'ouverture de ce généreux système de diffusion à un grand nombre de publications de divertissement. La crise de Presstalis nous a imposé de reconsidérer l'accessibilité, afin de mieux la recentrer sur l'intérêt général, donc sur la mission d'information de nos concitoyens, sans toutefois mettre en danger la presse spécialisée. Enfin, ce texte apporte une réponse aux préoccupations des kiosquiers et de leurs clients. Il s'agit d'un enjeu majeur dans les territoires tenus en marge de la transition numérique par les retards d'installation d'infrastructures.

s'étaient d'ailleurs attachés à ce que la garantie du pluralisme nécessaire à un débat d'idées équilibré figure désormais parmi les objectifs de l'Arcep. En effet, il nous paraît essentiel d'inclure cette préoccupation dans le logiciel du nouveau régulateur, afin qu'il puisse adapter ses pratiques dans ce nouveau champ de compétences qui s'offre à lui. Nous saluons donc le maintien de notre amendement. Nous nous réjouissons par ailleurs d'avoir été entendus quant aux modalités de saisine en urgence de l'Arcep en cas de manquement à l'obligation de distribution d'un titre de presse. À l'inverse, nous avons entendu les arguments concernant notre proposition, adoptée par le Sénat, de transformer l'avis simple des maires en avis conforme, en cas d'installation de points de presse en zone commerciale. Il s'agissait de permettre aux maires de protéger la vitalité de leurs centres-villes. Nous verrons à la longue s'il faut y revenir : nous n'y reviendrons pas pour l'instant. Il nous faudra encore veiller à la vitalité des titres de presse, point que nous avions souligné au moment des débats sur les conditions de diffusion des premiers numéros. Nous soutiendrons ce projet de loi. Mais, à l'heure de l'adopter, la faiblesse de notre droit s'agissant de la diffusion d'informations en ligne reste ma plus grande préoccupation. Peu de nos concitoyens le savent : les modalités d'acheminement de l'information sur internet échappent aux règles garantissant le pluralisme et les grands principes de la loi Bichet, y compris sur les sites internet de grands titres de presse. C'est la conséquence du modèle économique adopté par les acteurs du numérique, qui, en traitant toutes les informations comme des produits sans isoler l'information politique et générale, conduit à rendre les choix éditoriaux plus opaques et à enfermer le citoyen dans un algorithme de « préférences » sollicitées ou déduites de son activité en ligne, sur lequel nous n'avons que peu de prise

Tout d'abord, comme présidente de commission, je ne peux que souligner la très grande qualité du travail accompli par notre collègue Michel Laugier, qui était rapporteur pour la première fois. Il a su faire preuve, tout à la fois, de diplomatie et de fermeté pour faire valoir les convictions exprimées de longue date par le Sénat. Au-delà de cette réussite sur un sujet technique et- il faut bien le dire -très complexe, je suis heureuse de constater que notre commission, notamment dans le domaine de la presse, a su faire entendre sa voix et ses positions. Fortes

C'est dans nos territoires que bat le coeur de la presse nationale, de la presse locale, de la presse magazine, de la presse sportive, bref de toute la presse. Le système français de distribution, unique au monde, vise à créer les conditions d'une égalité entre nos concitoyens

préserve cette spécificité française d'une égalité dans la diffusion. C'est un premier point positif, et nous devons nous en réjouir, car des projets beaucoup plus durs auraient pu être présentés.

place résolument au centre de ses préoccupations ces marchands de presse trop longtemps ignorés. Le nouveau système, qui entrera en vigueur progressivement, permet d'envisager la fin de cette spirale mortifère de fermetures en créant les conditions d'une réelle autonomie des marchands. Ainsi, ces derniers pourront adapter beaucoup plus facilement leur offre de presse aux attentes de leur lectorat, bien entendu dans le respect de la diversité et du pluralisme. Disons-le franchement : nous espérons tous voir finir ce spectacle désolant de cartons entiers remplis de publications en nombre tel que les rayonnages croulent littéralement. Cette autonomie des marchands de presse, que toute la profession attendait, devrait- nous l'espérons sincèrement -permettre un sursaut et un surcroît d'attractivité pour cette profession, et et donc pour nos territoires. J'ajoute que, sur l'initiative de Michel Laugier, un avis du maire sera maintenant requis pour l'ouverture d'un point de presse. Cette disposition me semble de nature à permettre une meilleure association des maires au développement de ces commerces de proximité si particuliers.

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Personne

et à l'économie circulaire. Je vous indique également que, à la reprise de la séance, un moment de recueillement sera observé en hommage à Jacques Chirac, ancien président de la République, décédé ce matin. La séance est suspendue.